Elles prévoient le maintien chaque mercredi d'une séance de questions d'actualité au Gouvernement, sous le format adapté et restreint déjà mis en place, pour le restant des semaines du mois d'avril. En l'absence d'observations, je les considère comme adoptées.-

selon un sondage paru ce matin, 67 % des Français disent avoir bon moral, malgré la situation sanitaire et les mesures de confinement. Nous savons que le pic de la contagion est encore devant nous, même si la courbe s'est heureusement Cependant, nul ne peut nier que les conséquences économiques et sociales seront graves et nous affecteront fortement. À mon tour, je remercie toutes celles et tous ceux qui participent à l'effort national, notamment le personnel soignant, bien entendu, sans oublier les Français qui suivent les consignes de sécurité.

Tel est l'objectif du confinement. Pour faire face au nombre élevé des cas sévères, nous avons considérablement augmenté notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. J'y insiste, parce qu'il s'agit en

tout en continuant d'accueillir, dans des conditions de tension considérable, un nombre de malades en situation grave, souvent pendant une très longue période. C'est exceptionnel. La mobilisation du système de soins, c'est bien évidemment l'engagement des personnels soignants,

de fatigue qu'il faut évidemment bien avoir en tête. C'est la raison pour laquelle, je le dis régulièrement, l'heure du déconfinement n'est pas venue.

après maintenant plus de trois semaines de confinement, l'immense majorité de nos concitoyens a pris la mesure des règles de sécurité sanitaire à appliquer. Bien sûr, toutes ces contraintes sont difficiles à vivre. Je me réjouis de la vertu civique de tous ceux qui ont compris que nous vaincrons aussi ce virus par notre responsabilité collective. À charge, pour l'État, de transmettre des recommandations claires et cohérentes, qui seront ainsi d'autant plus efficaces.

Nous devons les protéger. Pour beaucoup de Français, aller faire ses courses est devenu la seule sortie, créant parfois un « effet promenade » irresponsable lorsque cette sortie devient familiale ou s'étire dans la durée. Si votre gouvernement a déjà restreint la tenue des marchés en lieux ouverts, aucune norme n'a encore été édictée pour préciser les conditions d'accueil du public dans les grandes surfaces et protéger les salariés comme les clients. Cette réglementation est pourtant indispensable, dès lors que les grandes surfaces captent l'essentiel de la distribution alimentaire et peuvent, en outre, vendre d'autres produits. Monsieur le Premier ministre, des propositions sont déjà sur la table. Par exemple, en Loire-Atlantique, un groupe de soutien scientifique créé sur l'initiative de notre collègue Ronan Dantec a formulé plusieurs recommandations,

Le pays a réussi à trouver une façon de garantir l'approvisionnement alimentaire, et je veux saluer tous ceux qui participent à cet effort, qu'ils soient producteurs, agriculteurs ou commerçants de la

C'est la raison pour laquelle la ministre du travail, avec les organisations syndicales et toute une série d'experts, a lancé une réflexion visant à produire des guides de bonnes pratiques, métier par métier, activité par activité. Ces documents sont très

des solidarités et de la santé, quand la pandémie a frappé notre pays, médecins et personnels soignants vous alertaient depuis des années. Vous refusiez de les écouter.

Mais ils ont la rage au coeur. Le dévouement n'a pas effacé la colère, monsieur le ministre, soyez-en sûr. Aujourd'hui, vos mots changent. Vous dites : « Rien ne sera plus comme avant ». Le Président de la République a affirmé, au fil de ses déclarations, que « la santé gratuite est un bien précieux », qu'« il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché » et qu'« un plan d'investissement massif devra être conduit pour l'hôpital public ». Que vont devenir ces mots, monsieur le ministre ? Nous apprenons par exemple avec stupéfaction, par, qu'une note d'experts de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), commandée par l'Élysée, prévoit au contraire d'aggraver la marchandisation de la santé et de l'hôpital. C'est hallucinant, alors même que dans le pays les balcons non seulement applaudissent, mais désormais se couvrent de banderoles pour demander- je cite, par exemple, les termes d'une pétition qui vient de recueillir 100 000 signatures en quelques jours -« de l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital » ! Monsieur le ministre, j'ai deux questions.

passe par une concertation. Il est indispensable que nous demandions à celles et à ceux qui font l'hôpital aujourd'hui, et qui sont applaudis par les Français, ce qu'ils attendent de l'hôpital, de leur outil de travail, pour aujourd'hui comme pour demain.

pas satisfaits par l'État. Des régions, des départements et des communes se sont démenés pour combler les manques, notamment en masques. Ils l'ont fait en informant l'État, par l'intermédiaire des préfets et des agences régionales de santé L'État a malheureusement pu donner l'impression de ne pas être capable d'accompagner l'action de chacun de ces acteurs. Un épisode malheureux a ainsi eu lieu lors de la réception d'une livraison de masques commandée par les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, ainsi que par l'État. En effet, l'armée a réquisitionné, sur le tarmac, l'ensemble de la commande. Cette réquisition aurait pu être comprise si elle avait été annoncée, expliquée ou justifiée. Il n'en a rien été ! Plusieurs autres cas similaires constatés sur le territoire national renvoient aux élus locaux un sentiment décourageant de frustration, voire d'inefficacité. Ceux qui voient les masques dont ils ont besoin partir vers d'autres territoires le ressentent même comme une expression de mépris à l'égard de leur propre population. Alors même que, sur le terrain, le dialogue est bon entre l'État territorial et les élus, comme entre les élus eux-mêmes, l'État central continuer de donner le sentiment qu'il improvise, faute d'avoir suffisamment anticipé, et qu'il coordonne mal ses troupes, préfets et ARS. Cette question de la confiance et de la coordination entre les acteurs est primordiale. Nos besoins en masques ne vont pas diminuer ; un nouveau changement de doctrine concernant le port des masques est d'ailleurs attendu. Monsieur le ministre, allez-vous transmettre et faire appliquer des consignes claires, pour que l'État régule, coordonne et ne parle que d'une seule voix vous posez la question des difficultés d'approvisionnement en masques

Dans le cas particulier que vous évoquez, il n'y a pas eu de réquisition, ni par l'armée ni par qui que ce soit. Il y a eu des commandes- des commandes légitimes, fortes, faites par des collectivités locales et par l'État, et en particulier par l'ARS du Grand Est. Cette dernière avait commandé et

cet importateur avait aussi pris les commandes de deux collectivités locales, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département des Bouches-du-Rhône. Au moment de la livraison, seuls 3,4 millions de masques étaient

du numérique, les Français confinés utilisent massivement le numérique pour travailler à distance, pour faire leurs achats, pour se divertir ou encore pour échanger avec leurs proches. La géolocalisation peut être par ailleurs un outil pour traquer les déplacements et endiguer la diffusion du Covid-19.

La situation actuelle révèle et renforce notre dépendance aux Gafam. Ces géants prennent une part de plus en plus prépondérante dans notre économie, sans payer d'impôts à la hauteur de leurs profits. Les entreprises françaises souffrent pendant que ces géants gagnent des parts de marché. Il serait normal que les entreprises qui, en définitive, bénéficient de cette crise contribuent financièrement à aider celles qui en pâtissent.

Nous devons penser cette crise comme une occasion de modifier notre modèle de développement, trop dépendant d'autres nations dans des domaines majeurs. Monsieur

ont massivement recours aux outils numériques des entreprises américaines. Même l'État, dès lors qu'il s'agit par exemple d'organiser des visioconférences, décide instantanément-

à la crise. Monsieur le Premier ministre, l'État n'est pas seul face au Covid-19. Tout d'abord, il y a tous les Français, sans lesquels le confinement ne pourrait être efficace- il faut d'ailleurs l'esprit de discipline dont, globalement, ils font preuve, ainsi que leur esprit de responsabilité individuelle dans l'intérêt collectif. Ensuite, il y a les collectivités territoriales les maires, qui assurent la continuité du service aux habitants, qui sont à l'écoute des plus vulnérables et qui fournissent aux écoliers le matériel dont ils ont besoin ; les départements, qui ont mis à la disposition de l'État les laboratoires départementaux et interdépartementaux, afin de réaliser les tests de dépistage, mais qui s'occupent aussi des collégiens et des personnes âgées ou handicapées ; les régions, qui participent au fonds de solidarité que vous avez mis en place. C'est toute une harmonie qu'il faut réussir à créer entre les différents

jeunes d'entre nous, de nos grands-parents âgés, en particulier ceux qui résident dans les maisons de retraite médicalisées. La commission des affaires sociales a entendu, ce matin, la présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous constatons que, dans de très nombreuses maisons de retraite, le personnel n'a toujours pas, en nombre suffisant, les masques dont il a besoin pour éviter les contaminations. Il est très important que le Gouvernement accélère la mise à disposition, pour ce personnel, des équipements qui sont indispensables, afin de faire face au risque d'épidémie mortifère dans les maisons de retraite. deux aspects dans votre question : le problème général de la collaboration entre l'État et les collectivités territoriales dans la gestion de cette crise sanitaire et la situation spécifique des personnes âgées en situation de dépendance et, plus généralement, de toutes les personnes fragiles accueillies dans des structures collectives. Je commence par le premier aspect de votre intervention. Vous avez raison de le dire, dans une crise sanitaire, il y a bien sûr l'État, mais il n'y a pas que lui : il y a la Nation, les collectivités territoriales et les entreprises. heureusement, depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons vu, à côté de l'État et souvent en bonne intelligence avec celui-ci, de très nombreuses autres entités,

les entreprises les plus petites qui se trouvent confrontées à une interruption, complète ou partielle, de leur activité, donc à une difficulté qui met en cause leur existence même.

à leur tâche, notamment à l'hôpital. Cette collaboration, nous entendons la chérir, la préserver et la développer. C'est la raison pour laquelle, lorsque je reçois les responsables je le fais avec les présidents des grandes associations d'élus, de sorte que chacune des strates importantes de collectivités territoriales soit informée et, dans toute la mesure du possible, associée. Pour ce qui concerne les personnes les plus fragiles accueillies dans des structures collectives,

Le ministre des solidarités et de la santé a indiqué que sa priorité était de développer les tests, notamment virologiques, dans les Ehpad et dans les structures collectives dont nous parlons. Pour le faire dans de bonnes conditions, il faut évidemment s'appuyer sur les laboratoires départementaux, que vous avez vous-même évoqués.

faire en sorte que cette intelligence des territoires, cette coordination des bonnes volontés et des compétences, puisse se faire dans les meilleures conditions. Je le sais, il y a çà et là des frottements et des différences d'approche ; ce n'est pas anormal et, au fond, cela ne nous surprend pas.

à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui débouchera sur une crise économique sans précédent. Dans leur grande marge majorité, les Français, anesthésiés par le confinement et par la peur du virus, mais la catastrophe économique à venir entraînera de graves conséquences sociales. Le Gouvernement a pris la mesure de la gravité de la situation, en lançant un premier plan de soutien économique : délais de paiement pour les charges sociales et fiscales, rééchelonnement des crédits bancaires, mobilisation de Bpifrance, simplification et renforcement Parmi les mesures les plus notables, figure la possibilité, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs de différer le paiement des charges sociales ou des impôts directs. Cette mesure a offert une respiration salutaire à ses bénéficiaires. Elle était nécessaire ; elle nous paraît aujourd'hui insuffisante. La perspective d'un décaissement important à venir de ces sommes est comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de structures dont la pérennité est menacée. Même avec des facilités de paiement, nombre d'entre elles ne pourront pas payer ces charges reportées, n'ayant perçu aucune recette pendant la période de confinement et ne disposant d'aucune réserve ou marge financière dans leur activité.

le cas, nous sommes bien conscients qu'un tel dispositif devrait être strictement encadré, pour éviter fraudes, abus et effets d'aubaine. Ainsi, quels pourraient être, selon vous, les critères à réunir pour bénéficier d'un dégrèvement de dette sociale et fiscale ? La parole

aux entreprises le demandant et remplissant les critères de bénéficier d'un crédit de trésorerie qui représente 25 % de leur chiffre d'affaires annuel.

secrétaire d'État, de nous avoir confirmé que le principe d'une annulation de charges, ciblée sur certaines activités et certaines structures, était envisagé par le Gouvernement. Nous comprenons que le cadre de cette éventuelle annulation reste à définir. Quels secteurs d'activité, quel type d'entreprise, quelle période prendre en compte ? Le Parlement et le Gouvernement pourraient envisager une réflexion commune pour définir ces critères. Comme toujours, le Sénat est prêt à contribuer à cette indispensable réflexion. La parole est à M. Philippe Pemezec, pour le groupe Les Républicains.

À défaut d'avoir su faire face aux premiers assauts de la guerre sanitaire, l'État aura au moins retenu la leçon économique et financière de la crise de 2008. Une aide forfaitaire et apparemment généreuse a été mise en place pour les TPE, les indépendants et les micro-entrepreneurs, le fonds de solidarité. Cette mesure est insuffisante : de nombreuses TPE devront malheureusement mettre la clé sous la porte. Imaginez un restaurateur sans chiffre d'affaires, qui doit payer ses factures et ses charges Les TPE, ne l'oublions pas, représentent 3,3 millions d'entreprises, soit 95 % du tissu économique. Elles emploient 20 % des salariés en France. Elles sont le coeur qui fait battre et respirer nos communes. Monsieur le Premier ministre, si les banques vous répondent encore, elles ne prennent plus au téléphone nos artisans ni nos commerçants. Et si elles les lâchent, ce sera un abîme dans la fracture territoriale.

Deuxièmement, quand utiliserez-vous tout votre poids pour faire pression sur les banques et les assureurs ? Je rappelle que les banques ont été sauvées par l'État, c'est-à-dire par le contribuable, lors de la crise de 2008. Ne serait-il pas normal qu'elles fassent à leur tour un effort ? Troisièmement, et enfin, vous avez affirmé à l'instant que les communes jouaient le jeu.

Pemezec, vous l'avez rappelé, nous sommes aux côtés des entreprises et nous n'avons pas attendu. L'État a fait montre de sa très grande réactivité, épaulé en cela par la représentation nationale, qui a très vite voté les mesures que nous lui avons proposées.

assureurs ont de surcroît accepté de repousser le paiement des primes sans remettre en cause l'intégrité des contrats. C'est un effort solidaire, manifeste

Je tenais tout d'abord à saluer le courage et l'engagement des personnels, qui, depuis le début de l'épidémie, sont allés travailler, parfois avec « la peur au ventre ». Trop longtemps, en effet, ils ont manqué des moyens de protection Alors que ces professionnels sont, depuis plusieurs années, confrontés à des difficultés structurelles, dues au manque de moyens financiers et humains, ils ont su trouver les ressources pour faire face de manière admirable à cette crise. J'espère sincèrement que, lorsque que, lorsque viendra « le jour d'après », on ne s'empressera pas de les oublier ! Vous avez annoncé le lundi 6 avril dernier le lancement d'une « vaste opération de dépistage » dans ces établissements. C'est une mesure que je salue : elle permettra de mieux gérer la situation. L'un des problèmes à traiter en priorité est celui de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je reprendrai les mots du psychiatre Michel Debout, professeur émérite de médecine légale, qui explique que la présence des membres de la famille dans les derniers instants d'un proche est tout à la fois « la condition psychologique, affective et émotionnelle, pour permettre à la personne âgée de mourir dans la sérénité » et la condition pour « la famille de ne pas ressentir qu'elle a abandonné une dernière fois son parent Il redoute ainsi que « beaucoup de ces familles ne présentent, une fois la crise sanitaire passée, des états de deuil pathologique, qui viendront pour une longue période dégrader leur vie psychique et relationnelle ». Se pose de la même manière la question de la prise en charge des soignants, au lendemain de la crise. au lendemain de la crise. Je voudrais aussi dire un mot des agents des services mortuaires, derniers maillons de la chaîne du soin. Ils doivent à ce titre pouvoir, comme tous les soignants, bénéficier de toutes les protections face au virus. Comme le souligne très justement le professeur Debout, « notre humaine condition se construit, depuis la nuit des temps, sur le fait que nous soyons la seule espèce vivante qui enterre ses morts ; cette place donnée aux morts permet de les relier aux vivants et de construire avec eux la chaîne ininterrompue de l'humanité

Monsieur le sénateur Jean-Claude Tissot, votre question traite de l'humanité avec laquelle on affronte la fin de vie dans des conditions déjà difficiles,

Le Gouvernement a très vite annoncé des mesures pour répondre à l'urgence de la situation, mais nous savons que ces violences faites aux femmes comme aux enfants sont aggravées par le confinement.

de se signaler depuis leur domicile. C'est pourquoi il convient que les forces de l'ordre, auxquelles nous tenons à rendre hommage, puissent assurer le suivi des mains courantes et des plaintes. Est-ce bien le cas ? À côté de l'État, les conseils départementaux jouent un rôle essentiel dans la protection de l'enfance et la lutte contre les violences faites aux femmes

Seule la fin du confinement dévoilera l'ampleur des violences intrafamiliales. Les services de protection l'anticipent-ils ? Dans l'immédiat, vous annonciez, avec Mme Schiappa, un million d'euros à destination des associations. Quels sont les critères d'attribution ?

notamment avec la livraison de trente téléphones portables. Nous avons déclenché le plan de continuité du 119, le numéro de l'enfance en danger. Aujourd'hui, une trentaine d'intervenants

Nous avons enfin, avec la garde des sceaux, assuré la permanence pour les audiences urgentes pour mineurs et la prise d'ordonnances de protection pour les femmes et les enfants quand c'est nécessaire, ainsi que le maintien des comparutions

de 1 million d'euros, répartie en trois grands volets : soutien à l'hébergement des femmes victimes de violences, soutien à l'hébergement des auteurs de violences conjugales et soutien à des associations nationales et de terrain.

Cette phrase a un mois, quasiment jour pour jour. Elle est du Président de la République, Emmanuel Macron, à propos de la crise du Covid-19. En une phrase, voilà résumées toute l'impréparation et l'incompétence de l'État, mais ce n'est pas une surprise. Depuis lors, nos compatriotes découvrent et subissent la litanie de vos mensonges, car vous avez menti, et vous saviez ! Vous saviez, depuis le 11 janvier dernier, quand Agnès Buzyn a prévenu le Président de la République et l'ensemble de votre gouvernement. Vous saviez, et vous avez choisi de mentir. Vous avez menti, et des Français sont morts. Le 18 février, le ministre de la santé, Olivier Véran, déclarait que la France était prête. Le 26 février, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, affirmait qu'il n'y avait pas de sujet de pénurie concernant les masques. Le 20 mars, c'est Laurent Nunez qui refusait de reconnaître le manque de masques. Mais alors, pourquoi Jérôme Salomon a-t-il affirmé, en privé, quatre jours plus tôt : « Les stocks de masques sont limités et on en cherche partout. ». Pourquoi, le 5 avril, Christophe Castaner a-t-il appelé les Français à donner leurs masques aux hôpitaux ? ? Le 13 mars, monsieur le Premier ministre, vous avez vous-même affirmé que porter un masque ne servait à rien. La réalité, c'est que vous avez menti sur les masques pour gagner du temps, sachant pertinemment que les stocks stratégiques avaient disparu depuis des années et que la France n'en avait plus. Conséquence : aujourd'hui, la préfète de la région Grand Est réquisitionne les 6 millions de masques destinés au personnel soignant des Bouches-du-Rhône et vous réquisitionnez les 4 millions de masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté. Cela vire à l'anarchie. Vous avez même réussi à faire voler en éclats l'unité nationale. Incapables de prévoir, vous êtes incapables de protéger la population. Si des Français sont en réanimation, n'en déplaise au sinistre préfet de police de Paris, c'est parce que votre gouvernement n'a pas su, pas pu ou pas voulu les protéger Tous ces drames, vous en êtes responsables. Et peut-être en serez-vous, demain, reconnus coupables. Voici ma question : pensez-vous, monsieur le Premier ministre, que vos mensonges successifs relèvent de la Cour de justice de la République ?